Le président Retailleau a tenté de faire valoir que des avis divergents traversaient nos travées. Tout de même

Le président Retailleau a parlé de « pari anthropologique », en reprenant l'expression de Jean-Pierre Chevènement, et dit que, au fond aucune étude n'avait permis de prouver quoi que ce soit ... Tout de même,

! Je ne veux pas que l'on nous fasse de leçon ! Au nom de M. Neuwirth et de Mme Veil, la droite n'a pas à recevoir de telles leçons de la gauche.

moment du vote de cet article 1, une question se pose : quel avenir pour les enfants privés de père ? Aucune étude d'impact sérieuse n'existe sur le sujet. Lors des auditions de la commission spéciale sur le projet de loi,

Au nom du principe de précaution, il ne faut donc pas voter cet article 1, car cette réforme anthropologique aura forcément des impacts psychologiques sur les enfants à naître sans père. Pour autant, je reconnais la diversité des familles françaises et la respecte. La

Je m'efforce de ne parler qu'au nom de la raison, de ma modeste raison, et dans le plus grand respect pour les conquêtes de la science.

Aujourd'hui, la science nous donne la possibilité d'artificialiser la conception et la naissance d'un être humain.

de vue de la raison, nous avons éthiquement le droit d'engager notre législation dans la voie de la reconnaissance de cette transformation très profonde de l'évolution de l'espèce humaine.

J'ai voté pour le mariage entre personnes de même sexe, parce que je croyais utile, voire nécessaire, de reconnaître socialement l'existence d'autres couples. Je ne crois pas, en

Ce qui est intéressant dans cette accusation de l'Académie nationale de médecine, c'est que l'on voit clairement qu'elle utilise un mot pour un autre. « L'Académie dit qu'il s'agit d'une rupture anthropologique comme s'il s'agissait de dire que la PMA sans père était contre nature Et comme on ne peut plus associer l'homosexualité et une supposée contre nature, l'Académie utilise cette périphrase : " rupture anthropologique ". « Mais précisément, le propre de l'anthropologie par rapport à une hypothétique nature humaine, c'est d'être constamment en mouvement. Toute l'oeuvre de Lévi-Strauss sur les systèmes de parenté vise à illustrer l'assertion selon laquelle il n'y a pas d'invariants humains, depuis les sociétés matrilinéaires jusqu'aux sociétés patrilinéaires, avec des communications incessantes entre les unes et les autres. La France a subi, par exemple, une rupture anthropologique au XIII siècle en matière de système d'héritage. Le Béarn a échappé à cette rupture, les Béarnais n'en sont pas moins humains et français »- enfin, je le crois.

préserve le naturel en la personne, puisque la nature, c'est aussi le désir de se prolonger, non pas le droit à l'enfant comme cela est dit souvent sur un mode péjoratif, mais le désir d'enfant qui semble être inscrit en la plupart d'entre nous. D'où cette question : au nom de quel système anthropologique une académie de médecine voudrait-elle interdire un désir aussi naturel chez l'humain que le désir d'enfant ? » La parole

développe usuellement cette pensée naturaliste, qui rejette la science et conduit à un certain nombre de positions non scientifiques. Évidemment, il y a des limites à poser,

ou moins heureux que les autres. Je veux dire surtout que, selon moi, le rôle de législateur n'est pas de décréter l'évolution des moeurs. Nous n'y pouvons rien, et qui serions-nous pour juger ?

entre l'ovule et le spermatozoïde : l'enfant n'est ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans la rencontre des deux. C'est un fait naturel ! Il nous appartient, parce que nous faisons société, de définir ce que sont la famille et le rôle des éducateurs,

Tout cela ne va pas changer grand-chose.

peut-être de droite, tout en étant un jour de gauche ou devenu progressiste. Non ! Je resterai à droite. explication de vote. En 1675, le Parlement de Paris interdisait la transfusion chez l'homme, sous peine de punitions corporelles. Encore maintenant, des sectes la refusent. Ainsi va le monde Aujourd'hui, la PMA est attendue en France par beaucoup. Elle est déjà autorisée dans plusieurs pays de l'Union européenne et accessible aux femmes qui peuvent passer les frontières.

suppression, car je souhaite que notre pays offre une nouvelle liberté, qui est attendue. Je ne me définis pas comme étant de droite ou de gauche, mais simplement comme un homme libre.

en ne me sentant ni de droite ni de gauche, mais simplement chargée de porter une loi qui traverse, me semble-t-il, tous les groupes parlementaires.

chaque technique médicale, pour savoir si elle met en tension un principe éthique fondamental. Or force est de constater que la PMA pour les femmes célibataires ou pour les couples de femmes ne met pas en tension nos principes éthiques fondamentaux. Elle peut choquer certains d'entre vous pour des raisons culturelles,

pourquoi. Cet article, tel qu'il doit être voté, ou pas d'ailleurs, ne met pas en tension des principes fondamentaux de nos lois de bioéthique, nos valeurs fondamentales, qui sont- je le répète -la non-marchandisation du corps humain, la dignité du corps humain le don altruiste. Et l'anonymat ! Ce sont aujourd'hui des raisons morales, culturelles ou religieuses qui fondent une position sur cet article, mais pas des raisons éthiques. Je ne porte pas

C'est bien parce que la France souhaite se doter d'un corpus éthique autour des questions scientifiques et médicales que nous avons ce moment démocratique, où nous discutons de ces nouvelles techniques et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre société. Les autres pays n'ont pas

il n'y a absolument aucune chance qu'une loi de bioéthique « à la française » puisse permettre cette façon de procéder que nous observons dans les autres pays, notamment européens.

aussi entendu le débat aujourd'hui, et l'on nous a tout de même expliqué que cet article 1, comme l'article 4 d'ailleurs, avait normalement sa place non pas dans une loi de bioéthique,

Je le dis d'autant plus fortement qu'il va falloir répondre à une autre question : celle de l'égalité. Aujourd'hui, vous ouvrez la PMA à des couples

vous avez affirmé que ce texte n'ouvrait pas un droit à l'enfant. Mais alors, vous devez pouvoir nous dire à quelles conditions l'on peut refuser l'accès à l'assistance médicale à la procréation d'une femme seule ou d'un couple de femmes.

en 1994. Ces lois réservent l'assistance médicale à la procréation aux cas d'infertilité médicalement constatés d'un couple formé d'un homme et d'une femme. Ce principe éthique a été reconduit successivement en 2004 et en 2011. Il s'agit donc de revenir sur un principe qui était jugé éthique. Il peut relever d'une opinion particulière de dire l'on ne remet pas en cause un principe éthique, mais vous me permettrez de considérer que, après trois débats parlementaires, ce principe constamment reconduit était bien un principe éthique. Enfin, pour aborder le fond du sujet,

dans la personnalité en formation d'un enfant qui devient adolescent, puis adulte, lorsque ce manque qui se creuse en lui ne trouve aucune réponse. C'est la raison pour laquelle je mets en garde contre la remise en cause de principes éthiques forts, que nous avons constamment soutenus et adoptés au Parlement. La parole est à Mme la ministre.

mettait en tension le principe éthique fondamental des lois de bioéthique française, c'est-à-dire la non-marchandisation du corps humain et la dignité du corps.

qu'elle soit pour une femme seule ou une femme en couple homosexuel, ne met pas plus en tension nos principes éthiques que la PMA pour des couples hétérosexuels. En réalité, la PMA aurait dû être ouverte depuis toujours aux couples homosexuels. C'est notre vision de la société qui a fait qu'elle n'a pas été autorisée, et non nos principes de bioéthique. Ce sont nos principes moraux ou la vision que nous avions de la famille. Au contraire, la GPA

Je rappelle que l'avis de la commission spéciale est défavorable, de même que celui du Gouvernement. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

qui ne vont plus être obligées de contourner la loi en allant quasi clandestinement en Espagne ou en Belgique pour avoir le droit d'être parents et d'élever un enfant.

de payer la PMA. Je voudrais citer l'une des phrases emblématiques de ce projet de loi : « Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs. »

D'un côté, on ouvre un droit ; de l'autre, on le réduit ... Notre amendement a pour objet de revenir à la rédaction issue de l'Assemblée nationale, qui ne souffrait, elle, aucune différenciation entre les couples pour une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale. Quel

Ce qui existe déjà, c'est la possibilité, pour les couples hétérosexuels infertiles, d'avoir recours à cette technique médicale qu'est l'AMP. Nous avons maintenu cette situation- autoriser le recours à l'AMP pour les couples hétérosexuels infertiles

où l'AMP pour les femmes seules et pour les couples de femmes n'est pas liée aux risques ou aux conséquences de la maladie, il n'y a aucune raison de la faire prendre en charge par la solidarité nationale. C'est une application assez logique du droit

ce qui nous concerne, nous voterons l'amendement présenté par Mme Cohen et ses collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Il s'agit de reprendre,

l'avortement, la fertilité et l'ensemble des activités sexuelles et reproductives. De ce point de vue, le remboursement de l'AMP pour l'ensemble des couples ou des femmes qui y postulent me paraît cohérent avec notre approche traditionnelle.

et l'autre pour les couples de femmes et les femmes non mariées. Vous pénalisez ainsi tant les couples hétérosexuels que les couples de femmes et les femmes non mariées. En effet, vous faites peser sur les premiers une condition, le maintien d'un critère médical, qui n'existera pas pour les secondes. Vous aboutissez donc à une inégalité que nous avons choisi d'éviter, d'autant que celle-ci aboutira forcément à des contentieux, qui obligeront à revenir à un régime identique pour tous.

aucune cause médicale ne peut être identifiée. La réintroduction d'un critère médical met en danger les réponses aujourd'hui apportées à ces couples. Pour ce qui concerne les couples de femmes et les femmes non mariées, l'instauration de deux régimes juridiques pourrait avoir pour conséquence pourrait avoir pour conséquence de ne pas rendre effectif le droit ouvert à ces nouveaux publics. En effet, ce double régime risquerait d'induire une priorité de prise en charge en faveur des couples hétérosexuels.

Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs. » L'adoption du présent amendement permettrait également de revenir au texte du Gouvernement pour ce qui concerne les limites d'âge pour de prévoir que ces limites soient fixées par décret en Conseil d'État, après avis de l'Agence de la biomédecine. Il existe aujourd'hui des arguments incontestables pour limiter l'âge du recours à l'assistance médicale à la procréation,

il est source d'inégalités et il fait l'objet de contentieux contre l'Agence de la biomédecine. Notre devoir est donc de poser des limites claires et de prévoir des bornes d'âge incontestables pour les équipes. Or la formulation retenue à l'issue des débats de la commission spéciale- « des conditions d'âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine » -ne me paraît pas de nature à répondre à ces exigences. Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite revenir au texte du Gouvernement : lever la condition d'infertilité pour tous les publics, reprendre le principe de non-discrimination dans l'accès à l'AMP et fixer des conditions d'âge d'accès à cette technique par décret.

de femmes et aux femmes non mariées dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels. Il s'agissait ainsi de ne pas faire de distinction selon l'orientation sexuelle ni le statut matrimonial des demandeurs. Or la commission spéciale est revenue sur cette extension harmonieuse, en conservant le critère pathologique pour l'accès des couples hétérosexuels à l'AMP. Mes chers collègues, au-delà des divergences que connaît notre assemblée sur ce sujet, force est de constater que, en pratique, cette position médiane soulève des questions. premier lieu, sur le plan de la logique juridique- j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, à propos d'un amendement que nous avons déposé -, le texte de la commission spéciale subordonne aux critères pathologiques la prise en charge de l'AMP par l'assurance maladie. Dès lors, comment justifier le maintien de ce critère pour les seuls couples hétérosexuels, alors qu'une femme seule ou en couple avec une autre femme peut présenter des problèmes d'infertilité entrant dans le même champ ? second lieu, le maintien de ce critère en lui-même, quels que soient les demandeurs concernés, ne semble pas aujourd'hui pertinent. Acceptons de regarder les faits : dans 15 % des cas, la mise en oeuvre de l'AMP ne s'inscrit pas dans un contexte pathologique. Comment justifier, en droit, le maintien d'un critère qui n'est déjà pas toujours appliqué dans la pratique ? Pour ces différentes raisons, guidés par un souci de cohérence, nous proposons de supprimer le critère pathologique pour l'accès à l'AMP des couples hétérosexuels.

pour être en conformité avec leur genre, mais cela pose un problème, qu'elles vivent extrêmement douloureusement : si une personne est née femme, mais change, quelques années plus tard, son état civil parce que son identité de genre est celle d'un homme, même si ses organes génitaux et reproductifs sont toujours ceux d'une femme,

qui s'est vu reconnaître le statut d'homme à l'état civil, tout en ayant conservé ses attributs féminins de naissance, n'est-elle pas à même de mener une grossesse à son terme ? Bien sûr que si, mes chers collègues ! L'état civil n'est tout au plus qu'un statut juridique. Souhaitez-vous véritablement créer une nouvelle inégalité de droits entre des personnes possédant les mêmes attributs génitaux et la même capacité à porter un enfant au simple regard d'une identité de genre ? J'espère bien que non. L'amendement n° 33 rectifié

n° 12 rectifié . Selon la philosophie de ce projet de loi, l'assistance médicale à la procréation est « la » solution en toutes circonstances et devient l'alpha et l'oméga de la lutte contre l'infertilité. Or le recours à l'AMP ne saurait être systématisé et banalisé tant il est loin d'être un long fleuve tranquille. Parcours douloureux pour la femme, il l'est aussi pour le couple, quand on sait qu'après les quatre tentatives de fécondation remboursées par la sécurité sociale, la moitié des couples reste sans enfant. Toutes méthodes confondues, le taux de succès des techniques d'AMP est de 17 %, et, en moyenne, il aura fallu concevoir dix-sept embryons pour une naissance. Dès lors, il est essentiel de poser comme principe que l'AMP ne peut être que l'ultime recours. Tel est l'objet de cet amendement.

Esther Benbassa et Laurence Cohen en ont parlé : toute personne en capacité de mener une grossesse, même en cas de changement de sexe à l'état civil, doit avoir accès à l'assistance médicale

La parole est à M. Henri Leroy. Il convient de réserver l'assistance médicale à la procréation aux couples formés d'un homme et d'une femme en cas d'infertilité dans un but thérapeutique, tout simplement.

Pourtant, la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU, ratifiée par la France en 1990, garantit le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, « de connaître ses parents et d'être élevé par eux

d'élargir la procréation aux femmes célibataires, au travers de ce projet de loi, et de créer des situations de vulnérabilité pour ces familles monoparentales et ces enfants à venir. Ne risque-t-on pas d'introduire une inégalité majeure entre les enfants, certains ayant,, un seul parent ?

et en autorisant le remboursement par la sécurité sociale pour des raisons d'infertilité, car 15 % de ces couples ne

insultant. Je le dis très clairement : les familles monoparentales ne sont pas à risque parce qu'elles sont monoparentales ; elles sont en difficulté parce qu'elles sont pauvres, plus pauvres que les autres. Leur vulnérabilité vient de leur pauvreté, de la pauvreté spécifique des femmes,

si vous discutez avec elles, elles vous diront que le pire, dans la monoparentalité, c'est la suspicion qui pèse sur leur capacité à assumer leur fonction parentale, à être de bonnes mères,

très malheureuses. Faire des généralisations à partir de son système de valeurs n'est pas un argument recevable. En l'espèce, laisser sa chance à chacun, y compris aux familles monoparentales, est

! Nous devons, dans cet hémicycle, être capables d'échanger des arguments. S'il est fait recours à des procédés d'intimidation, je demanderai une levée de séance.

ce n'est pas une raison suffisante pour vouloir créer de toutes pièces le même genre de situations par le fait du législateur, l'intervention du système de soins et le financement de la sécurité sociale !

nous avons examiné 34 amendements au cours de la journée ; il en reste 263 à examiner sur ce texte.